Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 26 mai prochain, les Français se rendront aux urnes pour élire leurs députés européens. Cette élection, nous en avons déterminé les règles l'année dernière, lors de l'examen de la loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen : une circonscription unique et une répartition proportionnelle des sièges français entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Ces principes, il n'est pas question de revenir dessus ; si nous nous retrouvons aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de notre fait, c'est parce que, depuis l'examen de ce texte, le contexte

le Brexit était initialement prévu pour le 29 mars dernier, c'est-à-dire deux mois avant les élections européennes. En conséquence, une partie des sièges britanniques au Parlement européen- vingt-sept des soixante-treize sièges, pour être précis

Néanmoins, vous le savez, les choses ne se sont pas passées, du côté britannique, comme prévu et les difficultés politiques internes de nos voisins ont poussé le Conseil européen à accorder un premier délai, puis un second courant jusqu'au 31 octobre 2019, pour permettre au Royaume-Uni de se mettre d'accord

Il nous fallait donc nous adapter, et le faire vite, pour permettre au scrutin qui aura lieu le 26 mai en France de se dérouler sans aucun risque, et dans les meilleures conditions possible.

en France ; c'est impératif pour assurer que ce scrutin puisse se dérouler sans aucun problème. Je sais que le Sénat a parfaitement pris conscience de la nécessité de traiter ce texte en responsabilité, et je veux sincèrement l'en remercier.

Enfin, je souhaite revenir sur un amendement du groupe du RDSE, qui a été déclaré irrecevable en commission, car il n'a pas trait au texte proprement dit, mais qui s'appuie sur des préoccupations que certains élus ont pu relayer, y compris auprès du ministre de l'intérieur.

mais le droit électoral doit néanmoins être respecté. Or je souhaitais indiquer que les panneaux électoraux sont justement conçus pour permettre de placer deux affiches côte à côte, et qu'il est donc d'ores et déjà possible et légal, si c'est nécessaire, de diviser par deux le nombre de panneaux électoraux devant les bureaux de vote. vote. Vous le voyez, tout doit être mis en oeuvre pour que les élections européennes se passent au mieux. Il est donc nécessaire de répondre à cette préoccupation des maires, tout comme il est nécessaire et urgent de tirer les conséquences des changements liés au Brexit. Tel est l'objet précis du texte que nous allons examiner

c'est-à-dire le jour où le Royaume-Uni cessera juridiquement d'être membre de l'Union européenne, où il ne sera plus lié par les traités qui régissent

cette décision européenne. Nous ne voyions pas de divergence, mais nous souhaitions que la rédaction du texte soit la plus claire possible.

pour la motion. L'article 14 du traité sur l'Union européenne, dit « traité de Lisbonne », définit le cadre de la répartition des sièges de députés européens entre les États membres : « Le Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges. « Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa. » En application de cet article 14, une décision du Conseil européen du 28 juin 2013 a fixé le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre pour la législature 2014-2019. Toutefois, cette décision viole de manière flagrante le principe de proportionnalité dégressive prévu par cet article, ce qui pénalise la France et, dans une moindre mesure, plusieurs autres pays.

La répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les nombres minimaux et maximaux fixés par le traité sur l'Union européenne afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres. d'autre part, le principe de la proportionnalité dégressive : « Le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l'arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et, à l'inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé.

avec les principes sus-évoqués, affirmés par le Conseil européen lui-même. En effet, en application de la proportionnalité dégressive, la France, qui est moins peuplée que l'Allemagne, devait également avoir un ratio moins élevé d'habitants par siège. C'est pourtant le contraire qui a été décidé, puisque ce ratio était de 852 539 habitants pour l'Allemagne et de 883 756 habitants pour la France. Lors de la préparation des élections de 2019, le Parlement européen a transmis au Conseil européen ses propositions de nouvelle répartition des sièges. À cette occasion, le Parlement a reconnu que « la répartition actuelle des sièges ne respecte pas le principe de proportionnalité dégressive à plusieurs égards et qu'elle doit donc être modifiée en vue de la composition du Parlement européen après les prochaines élections européennes, en 2019 ». La résolution du Parlement

Finalement, par une décision du 28 juin 2018, le Conseil européen a fixé la nouvelle répartition des sièges. Cette décision réduit de sept cent cinquante et des soixante-treize sièges britanniques, les vingt-sept autres sièges étant répartis entre quatorze pays de l'Union européenne pour compenser leur sous-représentation. En particulier, la France obtient cinq sièges supplémentaires, ce qui permet de respecter l'article 14 du traité de Lisbonne, puisque, dorénavant, le ratio d'habitants par siège serait, tenant compte des chiffres actualisés de population, de 854 838 pour l'Allemagne et de 843 818 pour la France. Toutefois, ce correctif était fragile, puisque la décision du Conseil prévoyait aussi le cas où le Royaume-Uni serait encore membre de l'Union européenne au moment des élections de 2019. Dans cette hypothèse, la répartition des sièges entre les États devait rester la même que celle qui a été utilisée lors des élections de 2014. Dans la mesure où la décision du Conseil européen du 28 juin 2018 devait être adoptée à l'unanimité des pays membres, il est donc clair que le gouvernement français a sciemment accepté une autre option, par laquelle, en cas de retard ou d'abandon du Brexit, en violation du traité de Lisbonne, notre pays n'obtiendrait pas le nombre de sièges qu'il devrait avoir au sein du Parlement européen.

Si ceux qui essaient de torpiller le Brexit parvenaient à leurs fins, cette injustice subsisterait. En effet, lors du Conseil européen du [28] juin 2018, la France a accepté que, en cas d'abandon du Brexit, la répartition actuelle des sièges soit maintenue à notre détriment, et ce en violation du traité de Lisbonne. » La ministre m'a répondu en m'accusant de diffuser des informations inexactes : « Nous Nous avons obtenu, contrairement aux informations qui vous ont été communiquées et qui sont inexactes, de rattraper ce qu'un mandat précédent n'avait pas su défendre, c'est-à-dire le nombre de députés européens auquel la France a droit. » Vous le savez, j'ai de la suite dans les idées ; j'ai alors posé la question écrite suivante à Mme Loiseau : le « Conseil européen a décidé que si le Brexit ne se concrétisait pas, la répartition des sièges entre les États resterait inchangée par rapport à la législature précédente. Dans cette hypothèse, la France continuerait à être victime d'une violation flagrante du traité de Lisbonne. La Constitution prévoyant que les traités internationaux doivent être respectés, » je lui demandais « s'il serait alors encore légal d'organiser en France des élections européennes sur cette base.

poli. Selon elle : « En tout état de cause, si le Royaume-Uni renonçait à sa demande de retrait, la décision du Conseil européen du 28 juin 2018 deviendrait caduque »- c'est totalement faux -, « obligeant ainsi ledit Conseil européen à adopter une nouvelle décision ayant pour objet de fixer la composition du Parlement européen pour la prochaine législature. C'est faux, je le disais, et, lors de la séance du Sénat du 14 février 2019, j'ai donc de nouveau effectué un recadrage en indiquant : « la décision [du Conseil européen] du 28 juin 2018 a prévu que, si le Royaume-Uni était toujours membre de l'Union européenne au moment des élections, l'ancienne répartition des sièges continuerait à s'appliquer jusqu'au départ effectif du Royaume-Uni. Dans ces conditions, si le Royaume-Uni partait dans six mois, dans un an ou dans dix ans, » voire ne partait pas, « on serait dans une situation évidente de violation du traité de Lisbonne ». Je continuais en m'adressant ainsi à la ministre : « Madame le ministre, je vous ai interrogée sur cette problématique par une question écrite n° 7142 au mois de novembre 2018. Vous m'avez répondu : " si le Royaume-Uni renonçait à sa demande de retrait, la décision du Conseil du 28 juin 2018 deviendrait caduque ". Madame le ministre, c'est de l'enfumage total et un mensonge à un double titre. Tout d'abord, rien n'indique dans la décision du Conseil du 28 juin 2018 que celle-ci deviendrait caduque en cas d'abandon du Brexit. Par ailleurs, les négociations avec le Royaume-Uni peuvent s'éterniser et durer pendant un an, deux ans ou plus : pendant toute cette période, nous continuerions à être dans une situation de violation du traité de Lisbonne. » Eh bien, mes chers collègues, comme je le pressentais depuis plusieurs mois, nous sommes bel et bien dans une situation de violation du traité de Lisbonne, et nul ne sait si le Brexit aura lieu. Le 26 janvier 2018, la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a adopté un rapport sur la répartition des sièges entre les États membres. En annexe, ce rapport comporte, pour chaque pays, les ratios officiels, pour l'Union européenne, d'habitants par siège dans les deux hypothèses- avec ou sans Brexit. On constate donc que, en l'absence de Brexit ou en attendant que celui-ci se produise, l'Allemagne, pays le plus peuplé, a maintenant un ratio de 854 838 habitants par siège est, pour la France, compte tenu de l'évolution démographique, de 900 833 habitants par siège et, pour le Royaume-Uni, accessoirement, de 895 085. La violation du principe de représentation proportionnelle dégressive est ainsi flagrante, au détriment de la France et, dans une moindre mesure, du Royaume-Uni. Étant le pays le plus peuplé, l'Allemagne aurait dû avoir un ratio d'habitants par siège supérieur à celui de la France ; ce n'est pas le cas, ce qui constitue une violation flagrante du traité de Lisbonne. Comme chacun le sait, la Constitution donne la priorité aux traités internationaux en vigueur sur les lois nationales. Dans la mesure où le projet de loi que nous examinons entérine la violation de l'article 14 du traité de Lisbonne, il n'est manifestement pas conforme à la Constitution

le Sénat interrompe sa discussion.

Par le passé, le financement des campagnes électorales était pour le moins opaque. Aux alentours de 1990, plusieurs affaires judiciaires ont été à l'origine d'une réglementation qui a plafonné les dépenses électorales, qui a, surtout, interdit les dons de personnes morales. En contrepartie, l'État a pris en charge les dépenses engagées par les candidats jusqu'à la moitié du plafond autorisé. Pour les élections où le plafond de dépenses est élevé- élections présidentielle, européennes ou régionales le système atteint toutefois ses limites, car les candidats doivent avancer des sommes considérables, et ils ne sont remboursés que plus de six mois après l'élection en question. De ce fait, ils sont obligés de souscrire des emprunts auprès des banques. Or on constate que, selon leurs affinités politiques, les banques pratiquent une discrimination entre les candidats. En général, elles accueillent avec beaucoup de bienveillance les demandes d'emprunt formulées par les partis dits « bien-pensants » ; au contraire, les partis qui contestent le système dominant sont, eux, victimes d'un ostracisme systématique. Lors de l'élection présidentielle de 2017, le Front national avait ainsi été obligé de souscrire un prêt auprès d'une banque étrangère, car les banques françaises lui refusaient tout financement. En matière électorale, l'argent est le nerf de la guerre et un parti qui est privé de moyens financiers pour faire campagne, subit un handicap rédhibitoire. Si une banque accorde un prêt à un candidat et le refuse à d'autres, le bénéficiaire profite, à l'évidence, d'un avantage en nature par rapport à ses concurrents. concurrents. Or un tel avantage accordé par une personne morale est interdit. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP, est très vigilante dans certains domaines. Par exemple, lorsqu'un candidat bénéficie gratuitement d'une salle municipale pour tenir une réunion, la CNCCFP exige la preuve que les autres candidats sont traités sur un pied d'égalité ; à défaut, elle pénalise le compte de campagne du bénéficiaire de la salle. une location de salle correspond à un avantage insignifiant par rapport à un prêt bancaire, lequel peut s'élever à plusieurs millions d'euros pour une élection nationale. Il est donc vraiment regrettable que la CNCCFP, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État n'aient pour l'instant pas réagi à l'encontre des discriminations pratiquées par les banques. Le problème est incontestable et il faut rendre hommage à François Bayrou, l'éphémère garde des sceaux du premier gouvernement d'Édouard Philippe, d'avoir évoqué le problème en proposant la création d'une banque de la démocratie. Malheureusement, les partis politiques dominants sont également ceux qui profitent du système, car leurs réseaux d'influence leur permettent d'obtenir des prêts sans grande difficulté.

À la place, ils ont créé un ectoplasme, à savoir le médiateur du crédit. En effet, non seulement ce dernier a une efficacité totalement nulle, mais il nie l'existence de tout problème et justifie les discriminations pratiquées par les banques. Lors des élections européennes de 2019, certains candidats ont été de nouveau confrontés aux mêmes difficultés que lors de la présidentielle de 2017. En l'espèce, le remboursement forfaitaire maximal de l'État est de 4,37 millions d'euros pour les listes atteignant le seuil requis de 3 % des suffrages exprimés. Les listes ayant, selon des sondages constants, la quasi-certitude de dépasser ce seuil auraient donc dû pouvoir emprunter sans problème auprès des banques. Pourtant, dès le début de la campagne, la presse a évoqué l'impossibilité pour certains partis politiques de souscrire des emprunts auprès des banques. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les exemples les plus cités sont ceux de partis qui contestent la pensée dominante : l'un à l'extrême droite, le Rassemblement national, ou RN, l'autre à l'extrême gauche, La France insoumise, est d'autant plus inacceptable que tous les sondages donnent la liste du Rassemblement national en première ou en deuxième position, avec plus de 20 % des suffrages. Ils donnent également la liste LFI aux environs de 9 %, soit trois fois plus que le seuil requis pour le remboursement.

De son côté, dans le même journal, un membre de la liste LFI indique : « Ce n'est pas aux banques de décider quelles sont les bonnes idées et quelles sont les mauvaises. C'est au peuple français de se prononcer. »

Il y a un certain nombre de critères à respecter. Celui de la solvabilité ne pose pas problème pour le Rassemblement national. Celui de la conformité, de la réputation et de l'image, c'est une autre chose. c'est une autre chose. » Ce pseudo-médiateur du crédit trouve donc normal qu'une banque défavorise un candidat en fonction de sa réputation au sein des pseudo-élites du microcosme politique. À mon avis, c'est scandaleux. Dans un article du 6 avril 2019, le journal a relancé le débat sous le titre « Européennes : les partis peinent à financer leur campagne ».

Des partis sans financement public parce qu'ils n'ont pas de parlementaires, avec peu de ressources et peu de garanties de franchir le seuil des 3 %, se posent en victimes. Mais les banques ne peuvent pas financer une activité à fonds perdu dès le départ. Ce serait quasiment du don. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout ce qui est pratiqué. À l'évidence, ce directeur aurait mieux fait de se taire, puisque le Rassemblement national remplit toutes les conditions énoncées : il bénéficie d'un financement public, il a des parlementaires et tous les sondages indiquent qu'il va pulvériser le seuil de 3 %. C'est bien la preuve du double langage du système bancaire. bancaire. Dans le même article, le médiateur du crédit réagit, une nouvelle fois, en totale contradiction avec sa mission. En effet, à l'égard des candidats victimes des banques, il propose une solution pour le moins surprenante : « Il n'est pas anormal de faire appel aux militants pour financer une campagne, les partis sont aussi faits pour ça. » Ainsi, selon lui, i1 y aurait deux catégories de candidats : d'une part, ceux qui ont le soutien des banques et qui, avec leur aide, peuvent financer sans problème leur campagne ; d'autre part, les victimes des banques qui n'ont qu'à se débrouiller, soit en faisant appel aux militants afin de rassembler les 4,37 millions d'euros correspondant au futur remboursement par l'État, soit en faisant campagne avec un handicap considérable par rapport à ceux qui sont aidés par les banques.

Il est donc absolument indispensable de garantir l'égalité de traitement entre candidats en créant une obligation pour les organismes bancaires d'accorder les mêmes conditions à tous les candidats. À défaut, il faut que le candidat ayant bénéficié des conditions les plus favorables soit réputé avoir reçu un avantage en nature de la part d'une personne morale. Le candidat et l'organisme bancaire seraient alors passibles des sanctions prévues pour la violation de l'article L. 52-8 du code électoral. Je regrette vivement

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, Brexit saison 2 ! Vous avez aimé la saison 1, qui s'est achevée le 29 mars ? Quel suspense, quel épilogue ! Combien d'heures passées à nous réunir pour analyser les échanges quotidiens au Parlement britannique, commenter les propos des et, voter des voter des textes pour nous préparer à l'apocalyptique scénario d'une sortie sans accord dont les parlementaires britanniques avaient pourtant clairement rejeté la perspective. Tout ça pour ça Nous voilà donc dans la saison 2 du Brexit, avec une nouvelle échéance fixée au 31 octobre prochain. Theresa refusait de discuter avec David durant la saison 1. Désormais, elle tente de le séduire. Elle lui propose de rester dans une union douanière temporaire jusqu'aux prochaines élections générales afin de créer une majorité pour concrétiser son Brexit. Mais David hésite. Et voilà une nouvelle échéance dépassée en avril. Le Brexit n'a pas eu lieu. Le Royaume-Uni fait toujours partie de l'Union européenne et les Britanniques sont contraints de convoquer des élections européennes. Coup de théâtre ! Ils participeront au renouvellement du Parlement européen qui interviendra dans dix jours. Si c'est une surprise pour certains, je voudrais leur rappeler que nous avions souligné, en avril 2018, que le Parlement britannique avait voté les crédits budgétaires pour participer aux élections européennes l'année suivante. Au risque de me répéter, je rappelle ce que j'ai déjà dit en juillet dernier : « En réalité, l'intérêt supérieur du Royaume-Uni n'est pas de quitter l'Union européenne. D'ailleurs, Theresa May préserve cette option. Lors du dernier conseil européen [de juin 2018], elle a remis une lettre destinée à permettre à son pays de participer aux élections européennes de 2019, si le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union européenne à l'échéance prévue. Voilà pourquoi, aujourd'hui plus encore qu'en juin 2016, moi qui vis au Royaume-Uni depuis plus de vingt ans, je reste convaincu que le Brexit n'aura pas lieu. Je n'ai pas changé d'avis depuis. Nous nous apprêtons à examiner un texte particulier. Alors qu'une partie des sièges des eurodéputés britanniques avaient déjà été répartis entre d'autres États membres, dont la France, nous voilà contraints de revenir sur cette décision pour le moins hâtive. Tel est l'objet de ce projet de loi que nous ne pouvons, bien évidemment, que soutenir. Dans dix jours, cinq candidats français seront entre deux eaux. Si les Britanniques restent dans l'Union européenne, ils ne siégeront pas. Theresa ne veut pas attendre le 30 octobre. Elle veut sortir avant le 30 juin pour que le Parlement européen nouvellement élu se réunisse sans les Britanniques. Je dois vous confier que la saison 2 lasse les gens. Les ressorts ne fonctionnent plus aussi bien. Le suspense s'essouffle. Personne ne croit, au Royaume-Uni, que la Première ministre britannique pourra convaincre son Parlement, le 4 juin prochain, de voter le texte qu'il n'a pas voulu adopter lors de la saison 1. Contrairement aux ordonnances que nous avons votées en début d'année pour amortir les effets d'une sortie sans accord du Royaume-Uni, il y a de fortes chances que le texte que nous votons aujourd'hui soit utile. Le Royaume-Uni est désormais profondément divisé. Une mauvaise ambiance s'est installée. Si le suspense s'estompe, la pagaille persiste. Les Européens qui vivent outre-Manche ont été invités à s'inscrire pour participer aux élections européennes en votant pour des listes britanniques. Il leur faut alors renvoyer par courrier postal un formulaire d'inscription sans qu'ils reçoivent d'accusé de réception. Pour surmonter cet obstacle administratif, deux ONG ont mis en place une procédure en ligne afin de faciliter la participation des Européens. Leur action a été stoppée par les autorités britanniques. Derrière le discours officiel, qui garantit aux citoyens européens le maintien de leurs droits existants, se cachent des faits, des chiffres révélés cette semaine

Ces données proviennent d'un rapport ayant fuité du et qui prévoit de restreindre significativement l'immigration d'Européens sur l'île dès la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. À la suite de cet article, j'aurais été heureux de lire une réaction de la France pour savoir comment le Gouvernement britannique justifie ses actions, alors que le droit européen est toujours applicable au Royaume-Uni.

Je vous l'ai dit, le climat n'est pas bon, et cela se ressent à la lecture des premiers sondages. Nigel Farage, celui qui a juré de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, puis de détruire l'Union européenne, caracolerait en tête.

Mais M. Farage est tout sauf un idéaliste. Il fait partie de la catégorie des nationalistes cyniques : prompt à dénoncer, invisible pour proposer C'est donc pour ce personnage, et pour quelques-uns de ses amis, que nous devons prévoir de faire de la place. S'il est bien une évidence qui s'impose devant le spectacle qui nous est infligé depuis bientôt trois ans,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « les institutions peuvent, si elles sont bien construites, accumuler et transmettre la sagesse des générations successives » : tels étaient les propos de Jean Monnet. Au moment où la campagne européenne est lancée et les candidats connus, il est important de rappeler les apports considérables, mais aussi les limites, d'une institution trop méconnue et politiquement sous-estimée. En effet, le Parlement européen, élu au suffrage universel direct depuis quarante ans, n'a cessé, au fil des années, de s'affirmer et de prendre du poids face aux autres institutions et particulièrement face aux États membres. Il est devenu le lieu d'expression démocratique de l'Union européenne et ses pouvoirs se sont renforcés progressivement : il est maintenant colégislateur dans quatre-vingt-cinq domaines de compétence allant du marché intérieur à l'environnement, en passant par l'énergie, les transports ou la politique agricole. Le Parlement européen est plus puissant que beaucoup de parlements nationaux et est indépendant de l'exécutif. Il dispose également d'un pouvoir budgétaire non négligeable, même s'il demeure sans compétence sur les recettes. C'est aussi lui, une fois installé, qui investit la Commission européenne et qui auditionne les commissaires européens avant leur prise de fonction officielle. Cela serait inimaginable en France. Entre 2014 et 2018, plus de 2 100 textes ont été adoptés, dont 708 textes législatifs. Et même si la quantité n'est pas gage de qualité, cela démontre indéniablement le dynamisme et le rôle prépondérant Il est souvent précurseur pour faire avancer des dossiers importants comme le paquet climat-énergie, les droits d'auteur ou le règlement général sur la protection des données, avec des positions beaucoup plus ambitieuses que les États. C'est aussi une assemblée qui protège les citoyens, comme ce fut le cas lors de la révision de la directive sur les travailleurs détachés ou sur la mise en place d'instruments de défense commerciale pour faire face aux distorsions de concurrence. Pourtant, et on peut le regretter, trop peu de nos concitoyens ont conscience du poids croissant du Parlement européen et trop peu s'intéressent au choix des députés européens, alors même qu'ils doivent traiter d'enjeux fondamentaux. Le taux Le taux très élevé d'abstention en Europe et en France- environ 60 % -, notamment chez les plus jeunes- trois sur quatre -, doit nous interroger. Il y a pourtant du choix pour les 41 millions d'électeurs français qui sont appelés aux urnes le 26 mai prochain avec 34 listes de 79 candidats officiellement enregistrées. Pourquoi ce Parlement européen reste-t-il si méconnu, quand il n'est pas parfois considéré comme illégitime ? Faut-il y voir une défiance des citoyens européens ? Le système électoral appliqué est-il pertinent ? Les causes sont multiples et interdépendantes crise générale de la démocratie représentative, pouvoirs proprement politiques de l'Union insuffisants, image lointaine, complexe et technocrate de l'Europe collant à la peau du Parlement, manque de relais locaux et nationaux, absence de pouvoir d'initiative parlementaire Et finalement, alors que les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis la semaine dernière, à Sibiu, pour parler, sans le Royaume-Uni, de l'avenir de l'Europe et des grandes priorités européennes pour les années à venir, l'ombre du Brexit continue de planer sur les élections européennes et sur l'Europe.

Selon un récent sondage, le parti de l'eurosceptique Nigel Farage est crédité de 34 % des intentions de vote, loin devant le parti travailliste, en deuxième position avec 21 %, soit une majorité d'eurosceptiques qui pourraient être tentés de perturber le travail et le bon fonctionnement du Parlement européen. Ce report du Brexit emporte également des conséquences directes sur les treize États membres qui se voyaient attribuer des représentants supplémentaires, mais qui vont devoir patienter et prévoir des règles transitoires. La France, qui devait gagner cinq sièges supplémentaires, compte tenu de son évolution démographique, passant ainsi de 74 à 79 représentants, a dû préparer ce projet de loi pour sécuriser et clarifier leur statut en précisant la méthode et le mode de leur désignation. Ce report compromet le renforcement de sa présence dans l'hémicycle européen et la prise en compte de l'évolution démographique de notre pays. On ne peut que le regretter. L'influence française s'en trouvera sûrement affaiblie, même si elle dépend aussi beaucoup de la présence de nos futurs eurodéputés français et de leur implication dans les différentes instances du Parlement européen. Espérons qu'ils auront à coeur de s'impliquer pour faire entendre la voix de la France. La complexité du fonctionnement des institutions européennes, la longueur et la difficulté d'approche des traités institutionnels, ainsi que la sous-médiatisation des enjeux communautaires, rendent difficile la démocratie européenne, même si nous ne devons pas oublier que l'Union européenne est garante de la paix en Europe depuis plus soixante Ce déficit démocratique est un problème. Une réflexion de fond s'impose aux citoyens européens et à nos dirigeants actuels et futurs. Le Parlement européen doit être une institution dynamique et un pilier de cette démocratie européenne. Les modalités d'élection des députés européens, qui ont évolué au fil des campagnes électorales, doivent être aussi une piste d'action à l'avenir pour renforcer la légitimité de l'Union européenne. Le groupe Les Indépendants soutient ce projet de loi. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, dans une tribune publiée le 16 mars dernier, Theresa May affirmait : « L'idée que les Britanniques se rendent aux urnes pour élire des députés européens, trois ans après avoir voté pour quitter l'Union européenne, est à peine supportable. Il ne saurait y avoir de symbole plus fort de l'échec politique collectif du Parlement. » On ne peut être plus clair Deux mois après cette déclaration de la Première ministre britannique, l'échec politique contre lequel elle mettait en garde la Chambre des communes est pourtant bel et bien consommé et il est désormais acquis que nous assisterons, le 23 mai prochain, à l'organisation ubuesque d'élections européennes outre-Manche. En effet, malgré la voix dissonante, mais isolée, de la France, les chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Sept se sont entendus, le 10 avril dernier, pour reporter de nouveau le Brexit. Après l'échéance initiale du 29 mars, repoussée une première fois au 12 avril, c'est donc désormais le 31 octobre prochain, au plus tard, que le Royaume-Uni quittera finalement l'Union européenne. Si l'on peut naturellement se féliciter qu'un certain réalisme politique ait prévalu afin d'écarter provisoirement le spectre du scénario catastrophe d'un, la durée de cette prolongation ne peut, en revanche, nous satisfaire. D'une part, elle allonge de six mois les incertitudes liées au Brexit, ce qui est dommageable d'un point de vue tant économique, en empêchant les entreprises de prendre des décisions fondées sur un horizon clair, que politique, en détournant l'Union européenne d'une tâche ô combien plus urgente, celle de son indispensable refondation face aux nombreux défis qui se posent à elle. D'autre part, ce nouveau calendrier non seulement vient parasiter le déroulement d'élections européennes particulièrement décisives, mais il risque également de perturber le bon fonctionnement des institutions européennes au moment même où des décisions structurantes devront être prises. Certes, le Gouvernement britannique s'est engagé, d'ici au Brexit effectif, à faire preuve de coopération loyale, c'est-à-dire à s'abstenir de prises de position qui qui pourraient entraver l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne comme, par exemple, l'utilisation de son droit de veto pour bloquer l'adoption du cadre financier pluriannuel ou pour compliquer la désignation du prochain collège Toutefois, rien d'autre que cet engagement moral n'empêchera le Royaume-Uni de voter comme il l'entend au Conseil, car il en restera membre de plein droit. En outre, ce principe de coopération loyale ne s'appliquera en rien aux députés européens britanniques, et c'est là qu'est le problème. On peut sérieusement douter que derniers, et en particulier les élus du, la nouvelle formation créée par Nigel Farage donnée largement en tête des intentions de vote, se sentent liés par l'engagement de Mme May et qu'ils acceptent de s'y soumettre.

à participer pleinement aux travaux du Parlement européen, mais on ne peut que s'interroger sur le rôle et le type d'influence qu'ils pourraient y exercer, dans une institution où les réunions en « format article 50 » n'existent pas. Dès lors, si les dirigeants européens ont jusqu'ici fait preuve d'une grande patience vis-à-vis des atermoiements du Royaume-Uni, celle-ci ne saurait être sans limites. D'autant que la patience des électeurs britanniques semble, elle, avoir atteint les siennes. Leur exaspération s'est ainsi traduite lors des récentes élections locales par la lourde sanction qu'ils ont infligée aux deux grands partis traditionnels, qu'ils tiennent- à juste titre -pour responsables des blocages sur le Brexit. Espérons que cet avertissement incite Theresa May et Jeremy Corbyn à accélérer les discussions bipartisanes qu'ils conduisent actuellement et dont on se demande d'ailleurs pourquoi elles n'ont pas été lancées plus tôt.

Espérons que cet avertissement incite Theresa May et Jeremy Corbyn à accélérer les discussions sur ce point. Un accord majoritaire concernant la relation future entre Londres et le continent ouvrirait la voie à une ratification du traité de retrait par la Chambre des communes. Et si un tel dénouement ne permet pas d'éviter la tenue des élections européennes au Royaume-Uni, il n'est pas totalement interdit d'espérer qu'il puisse intervenir suffisamment tôt, c'est-à-dire d'ici à la mi-juin, pour que les élus britanniques n'aient jamais à siéger au Parlement européen, dont la séance inaugurale- je vous le rappelle -se tiendra le 2 juillet. Néanmoins, le contexte politique qui prévaut actuellement au Royaume-Uni vient modérer cet optimisme, tant il demeure marqué par une confusion et une conflictualité extrêmement fortes. Tout compromis solide sur le Brexit reste ainsi particulièrement difficile à atteindre. Le gouvernement britannique a bien proposé aux travaillistes une solution consistant en un « arrangement douanier » avec l'Union européenne et en un « alignement dynamique » des droits des travailleurs britanniques sur ceux de leurs homologues européens. Mais si un accord devait être scellé sur cette base entre Mme May et M. Corbyn, il serait inévitablement combattu à la fois par les conservateurs, qui y voient notamment la trahison de la promesse d'une politique commerciale autonome, mais aussi par les travaillistes, qui sont nombreux à militer en faveur d'un second référendum. À ce stade, tout porte donc à croire que le projet de loi que nous étudions aujourd'hui, et auquel le groupe Les Républicains apportera son soutien, sera bel et bien nécessaire.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à quelques jours de l'élection européenne, permettez-moi pour commencer de rappeler les propos tenus par le président Emmanuel Macron lors de son discours d'Athènes d'Athènes : « En 2005, une page s'est tournée et nous ne l'avons pas vu tout de suite. C'est que l'Europe ne peut plus avancer à part des peuples. Elle ne peut continuer son destin que si elle est choisie, voulue. » Quel fossé entre cette déclaration, dont nous partageons le constat, et ce qui se passe aujourd'hui ! Non seulement aucune conséquence n'est tirée de ce diagnostic dans les politiques menées, dont le cours libéral continue à marche forcée, mais que constatons-nous, une fois de plus, avec l'organisation des élections européennes ? L'incurie démocratique et la médiocre qualité du débat des élections européennes demeurent la règle. Nous pourrions certes appréhender le présent projet de loi comme un simple détail technique. Il est vrai que les circonstances du Brexit obligent juridiquement, mais également politiquement, à conserver des représentants britanniques au sein de l'assemblée européenne jusqu'à ce que le retrait du Royaume-Uni soit effectif et définitif. Nous ne nous opposerons donc pas au projet technique présenté. Pourtant, force est de constater que cette situation, qui nous conduit à revoir les conditions de l'élection de nos représentants européens sans que les électeurs français saisissent rien, est révélatrice d'une Union européenne à bout de souffle démocratiquement. Les dirigeants britanniques et européens se sont jusqu'à présent montrés incapables de mettre en oeuvre une sortie pérenne et organisée du Royaume-Uni, quoi qu'on en pense sur le fond. Le Brexit a été un terrible aveu d'échec, et l'un des nombreux signaux d'une distanciation toujours plus forte des peuples Le chaos politique s'aggrave au Royaume-Uni, où le dangereux Nigel Farage pourrait rafler la mise de cet incroyable imbroglio. Quant à l'Union européenne dans son ensemble, cet épisode, après d'autres, révèle à quel point les dirigeants de cette Europe conçue seulement pour les marchés ne savent jamais quoi faire quand des peuples émettent des votes contraires à leurs intentions. En vérité, rien n'est jamais prévu pour qu'il soit tenu compte du vote desdits peuples.

Le traitement politique des conditions de l'élection européenne est lui aussi révélateur de cette incurie démocratique. Cet événement devait être un grand moment de débat démocratique. Or rien n'est réellement fait pour mobiliser l'intérêt de nos concitoyens. Les conditions de cette élection ont d'ailleurs, depuis l'origine, fait débat. Je rappelle que la loi fixant les modalités de la première élection des parlementaires au suffrage universel direct, en 1977, fut le premier cas, dans notre histoire constitutionnelle, d'utilisation de l'article 49-3 de la Constitution dans un domaine lié à nos relations extérieures. La participation aux élections européennes risque, cette année encore, de dépasser tous les records d'abstention elle avait déjà baissé de 20 points, en 2014, par rapport à 1979. La déception profonde causée par les politiques menées, leur rejet désormais majoritaire dans toute l'Union et l'opacité des processus de décision en sont les causes fondamentales. Et puisque ce projet nous donne l'occasion de revenir sur les conditions d'organisation de la campagne électorale, je veux redire notre colère sur trois points qui conduisent directement à alimenter la situation que je viens de décrire, faite d'asphyxie démocratique et de méfiance populaire.

Je redis, par ailleurs, que la répartition du temps de parole, issue du projet de loi dont nous avions dénoncé ici les travers, est un véritable scandale. Non seulement l'égalité du temps de parole n'est plus qu'un rêve, mais la répartition prévue par la loi aboutit à une caricature. nous, mes chers collègues, pèse royalement sept secondes de temps de parole par candidat ; et que donne concrètement ce tripatouillage législatif voté ici sans broncher l'an dernier ? La République En Marche se voit attribuer un temps de diffusion des clips officiels supérieur à celui des listes communiste, France insoumise, Europe Écologie Les Verts et Génération.s réunies ! Le Front national se taille une part de lion, concentrant plus de temps d'antenne que Les Républicains et l'UDI réunis. Le Gouvernement souhaitait favoriser indûment la polarisation entre La République en marche et le Rassemblement national ; la loi a exaucé ses voeux. C'est un choix dangereux pour la démocratie et l'avenir de l'Union européenne. Enfin, mes chers collègues, permettez-nous, à nous qui défendons ici si souvent le service public de France Télévisions contre les attaques dont il est l'objet, d'élever une protestation sur la manière dont France 2 organise le débat entre les listes présentées. Une première fois mise en échec,

débat. Les journalistes de France 2 réalisent bien souvent- je le sais -un travail sérieux et instructif dans des conditions difficiles. Ce ne sont pas eux que je mets en cause. Mais j'invite la direction de France Télévisions à revoir sa copie pour accorder un traitement juste et équitable à l'ensemble des listes. ! Il est temps, pour l'avenir démocratique de l'Union européenne, que soient créées les conditions d'un choix équitable des Français, qui supportent de moins en moins qu'on les prive de leur libre jugement. La

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en apparence, ce projet de loi relève du simple pragmatisme ; il répond à un besoin très spécifique : préciser comment, à la date éventuelle de sortie du Royaume-Uni, les cinq sièges supplémentaires qu'obtiendrait alors la France seraient pourvus.

donc de ce débat pour vous demander, monsieur le secrétaire d'État, de bien nous préciser que, dès lors qu'une personne est inscrite sur la liste électorale consulaire, elle aura la possibilité de voter après avoir été informée des sanctions pénales

entre le 23 et le 26 mai prochain, l'ensemble des citoyens européens est appelé aux urnes pour désigner les membres du Parlement de Strasbourg. Cette année, ce renouvellement se déroulera dans un contexte de grande incertitude, à la suite des rejets successifs par le Parlement britannique des accords de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous avons bien conscience, en outre, que près de 40 000 citoyens britanniques inscrits sur les listes électorales en France se trouveront, le 26 mai, dans une situation très paradoxale, alors que le dénouement de ce feuilleton devrait intervenir d'ici le 31 octobre prochain, avec l'adoption d'un accord de sortie auquel nous continuons de croire. Le groupe du RDSE se félicite malgré tout que 330 000 citoyens de l'Union européenne résidant en France se soient inscrits pour pouvoir voter aux côtés de nos concitoyens, tandis que 1,35 million de Français prendront part au scrutin depuis l'étranger. C'est le signe que les citoyens européens s'emparent de toutes les modalités de vote mises en place pour accroître la représentativité de notre système électoral. Néanmoins, l'absence d'accord de sortie placera également les électeurs français dans une situation inédite. Selon la solution entérinée par le Conseil européen du 28 juin 2018, nos concitoyens, comme ceux des États membres restants, voteront par anticipation anticipation du retrait britannique pour cinq représentants supplémentaires, qui entreront en fonction après ce retrait. Dans l'intervalle, le Parlement européen pâtira d'une légitimité affaiblie. C'est pourquoi nous espérons que l'accord que Theresa May s'est engagée à négocier avant l'élection du président du Parlement européen et la désignation de la Commission sera adopté. Dans le cas contraire, les parlementaires britanniques fragiliseraient toutes les démocraties européennes, dans un contexte de montée des populismes. Cela paraît inconcevable quand on connaît l'influence du modèle britannique sur la démocratie dans le monde ! C'est sur la base de cette logique que nous avions soutenu la position du gouvernement français de refuser un nouvel ajournement des négociations jusqu'en 2020. Comme l'écrivait Musset dans un tout autre registre : « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. » Très bien ! Celle entre le Royaume-Uni et l'Union n'est ni l'un ni l'autre il ne faudrait pas que les Européens en subissent plus longtemps les conséquences ! C'est ce qu'ont rappelé en substance les vingt-sept chefs d'État et de gouvernement en adoptant la déclaration de Sibiu, la semaine dernière. Dans ce climat particulièrement confus, nous sommes favorables à l'adoption de règles claires, et donc à ce que la règle de désignation des eurodéputés supplémentaire reste la même que celle s'appliquant au reste de leurs collègues- c'est ce que prévoit le projet de loi non amendé. Nous l'avions déjà rappelé l'an dernier, au moment de l'adoption du projet de loi portant rétablissement d'une circonscription unique : aucun système électoral n'est parfait. S'agissant des temps de parole applicables dans les campagnes électorales, la recherche d'une meilleure représentativité, d'une part, et, d'autre part, la nécessité de préserver le pluralisme, difficiles à concilier, sont de nature à produire des débats sans fin.

Sans entrer dans les détails de ce débat, il me semble que l'allongement de la durée totale de la campagne serait la seule solution consensuelle pour atténuer les frustrations. Nous savons également que, au temps des réseaux sociaux, les campagnes, désormais, se jouent peut-être ailleurs, et que notre combat pour le pluralisme devrait se mener dorénavant sur ces nouveaux terrains d'échange et d'expression. Les membres du groupe du RDSE sont ainsi tout à fait favorables à ce que, à la suite du scandale de Cambridge Analytica et de la publication du rapport Mueller, le Gouvernement prenne des initiatives au niveau national et international pour protéger les utilisateurs français de ces réseaux sociaux de tentatives d'influence malveillante, qu'il semble enclin à faire. Il y a là une réflexion essentielle à mener au bénéfice de notre jeunesse, dont les techniques d'information diffèrent considérablement des nôtres. Alors que la campagne électorale a commencé lundi dernier, je voudrais également rappeler à nos concitoyens l'importance du rôle du Parlement européen sur les nombreuses matières relevant de la codécision avec le Conseil, lorsqu'il ne se prononce pas à l'unanimité. Beaucoup de ces thématiques recoupent celles du grand débat il s'agit donc d'un rendez-vous essentiel pour convertir les réflexions amorcées ces derniers mois en actions concrètes. Au sein du Parlement européen, nos représentants sont en nombre suffisant pour peser dans les débats, contrairement à ce que certains voudraient laisser entendre- on sait à qui profite l'abstention ! Après le retrait britannique, la France y restera la deuxième nation représentée, derrière l'Allemagne, et la nouvelle répartition portera la part des représentants français dans l'hémicycle européen de 9,8 % à 11,2 % des sièges. À chacun de donner à nos futurs représentants une légitimité à la hauteur des nombreux défis qui les attendent, en participant à ce scrutin crucial pour l'avenir de l'Europe ! Très bien

collègues, notre excellent rapporteur a défendu il y a quelques semaines, en commission des lois, dans le

en effet d'apprendre que, depuis quinze jours, les partis européens peuvent financer les campagnes électorales. C'est extrêmement dangereux, mes chers collègues. Vous savez très bien que les partis européens sont financés par les structures de lobbying et que, par exemple, un parti européen que je ne citerai pas est financé par Bayer-Monsanto pour défendre le glyphosate

On a encore et toujours une incertitude quant au calendrier de sortie. Il a été fixé au 31 octobre. Certes, au regard de l'imprécision juridique de la rédaction de l'article 50, on pourrait envisager, d'un point de vue technique et juridique, que les Britanniques retirent

il faudra que les désignations fassent l'objet d'équilibres savants : équilibres politiques, qui seront en grande partie définis à la suite des résultats des élections européennes et des alliances qui se seront constituées